madame la présidente,

La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du samedi 24 novembre 2018 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Georges Benedetti, qui fut sénateur du Gard de 1986 à 1988.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 Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, la nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2018 aura lieu mardi 27 novembre, à quatorze heures trente. Acte est donné de cette demande. Par ailleurs, la conférence des présidents réunie ce jour a décidé, en accord avec la commission des finances et le Gouvernement, de modifier l'organisation de la suite de l'examen du projet de loi de finances pour 2019. Les explications de vote et le vote par scrutin public sur la première partie du projet de loi de finances se tiendraient jeudi 29 novembre. Le délai limite d'inscription de parole pour ces explications de vote serait également reporté au mercredi 28 novembre, à En conséquence, l'examen des missions initialement prévues les mercredi 28 et jeudi 29 novembre serait reporté, respectivement, aux samedi 1 et dimanche 2 décembre. Les délais limites de dépôt des amendements, initialement prévus aujourd'hui, à onze heures, pour les missions examinées mercredi 28 novembre et le mardi 27, à onze heures, pour celles examinées le jeudi 29 seraient également reportés, respectivement, au jeudi 29 et au vendredi 30, à onze heures. Les délais de cosignature et d'inscription de parole dans la discussion organisée seraient également reportés au vendredi 30, à onze heures. Il n'y a pas d'opposition ? ... Il en est ainsi décidé.

Le mouvement des « gilets jaunes » fait remonter à la surface toute la souffrance d'une grande partie de notre peuple qui, des exclus socialement aux classes moyennes, subit l'austérité dictée par les dogmes libéraux.

Cette réalité, beaucoup ne voulaient pas la voir, beaucoup la maintenaient sous le boisseau. La « trajectoire », terme très technocratique utilisé par le Gouvernement, d'augmentation de la taxe sur le carburant a mis le feu aux poudres.

Ce qui émerge, c'est une contestation profonde du libéralisme, comme le soulignait une pancarte ce samedi sur laquelle était inscrite : « Vos profits nous bouffent la vie Les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE ont déposé, comme d'autres ici, un amendement de suppression de l'augmentation de la taxe sur le carburant, et ils se félicitent de la probable adoption de ces propositions.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des finances demande la priorité sur les amendements et articles dont je vais vous donner la liste, afin qu'ils soient examinés au début de cette séance et dans l'ordre suivant les amendements portant article additionnel après l'article 18, sauf l'amendement n° I-463 ; l'article 19 ; les amendements portant article additionnel après l'article 19,

l'article 19 ; l'amendement n° I-890 portant article additionnel après l'article 7 ; l'article 33 ; l'article 8 ; les amendements portant article additionnel après l'article 8, sauf les

Gremillet. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cet amendement a plusieurs objectifs, dont certains sont en lien direct avec l'article 19, même si la commission des finances a souhaité scinder la discussion en deux. Comme l'amendement n° I-166 proposé par la commission des finances, il vise d'abord à geler les taxes sur l'énergie à leur niveau de 2018 pour tenir compte de la hausse des cours mondiaux et ne pas asphyxier les Français et notre économie. C'est là l'essentiel. Mais il vise aussi à maintenir le taux réduit pour le gazole non routier, le GNR, dont la suppression pèserait trop lourdement sur les secteurs concernés, en particulier sur celui du BTP. C'est là une différence majeure avec la commission des finances qui, elle, propose d'accepter cette suppression, mais d'en compenser les effets pour les PME un mécanisme de remboursement à l'article 19. Deux autres amendements tendent, par ailleurs, à répercuter la charge dans les contrats en cours, l'un pour les grands groupes, l'autre pour les entreprises qui utilisent le GNR de façon « significative Ces propositions ne sont pas satisfaisantes. La première alourdirait la charge administrative des PME et pèserait chaque année sur leur trésorerie, sans d'ailleurs atténuer le choc en 2019. Les deux autres reviendraient à faire payer les clients, à commencer par les collectivités publiques en matière de travaux publics. C'est pourquoi la meilleure solution consiste à maintenir, purement et simplement, le taux réduit plutôt que d'imaginer des dispositifs de compensation complexes ou qui reporteraient la charge sur d'autres. Nous sommes d'ailleurs nombreux à défendre cette position, si j'en crois les nombreux amendements déposés à l'article 19 pour maintenir le taux réduit en général ou pour toute une série d'usages spécifiques. Tous ces amendements seraient satisfaits par l'adoption de l'amendement amendement vise, par ailleurs, à créer ou à renforcer plusieurs taux réduits au bénéfice des biocarburants. Enfin, et bien qu'il ait été déplacé avant l'article 19, cet amendement tend à préserver deux autres points positifs l'exonération de l'ensemble du transport fluvial hors navigation de plaisance privée ; le remplacement, d'ici à 2021, du remboursement dont bénéficiaient les agriculteurs par un taux super réduit direct, qui leur donnera un gain net de trésorerie. un gain net de trésorerie. Cet amendement est un message politique adressé à nos concitoyens et à nos entreprises : le Sénat doit être pour le gel des taxes, pour le maintien du taux réduit et pour le soutien aux carburants alternatifs. Seul cet amendement permettra d'atteindre ces trois objectifs.

de fixer à l'avance une trajectoire pluriannuelle d'augmentation de la TICPE, et ce pour deux raisons. Premier motif, cette trajectoire risquait- c'est malheureusement ce qui s'est produit -d'être déconnectée des cours de l'énergie puisque nous avons fixé jusqu'en 2022 une augmentation pluriannuelle sans avoir idée de l'évolution du marché. Le deuxième motif qui nous avait conduits à refuser cette trajectoire pluriannuelle était l'absence ou la faiblesse des mesures d'accompagnement.

qui a d'ailleurs mené nombre de nos compatriotes à s'équiper en véhicule à traction diesel, la démarche mise en oeuvre depuis plusieurs années a été de mettre en place une forme de « convergence » entre la taxation du gazole et celle des autres carburants. Sauf que, derrière les vertueux principes environnementaux affichés, figurait en arrière-plan la volonté de conduire une profonde transformation de notre fiscalité comme de nos prélèvements sociaux, éloignant toujours plus ceux-ci de la sphère de la production pour investir celle de la consommation et du revenu.

Voilà une bonne idée ! La TICPE devrait rapporter, en 2019, 37,7 milliards d'euros, dont 17 milliards iront dans les caisses de l'État, alors que l'impôt sur les sociétés va dégager 31,5 milliards d'euros.

sociétés ? On marche sur la tête ! Voilà pourquoi nous proposons, à travers notre amendement, de procéder à un alignement à la baisse des taxes sur les carburants. Il nous semble nécessaire de marquer un coup d'arrêt, dans un premier temps, dans la progression de ces taxes et de procéder ensuite à l'inscription d'une tendance baissière.

Elles appellent, au contraire, des choix politiques forts, déterminés, revenant par exemple sur la programmation des fermetures de lignes de train, sur le développement des transports collectifs, dans le respect des principes de service public- loi du contenu

et les énergies fossiles, ne laissant qu'une part infime de leurs capacités de financement au secteur des énergies renouvelables. La formule n'est peut-être pas nouvelle, mais je trouve que c'est un véritable scandale

tend à créer une nouvelle ligne fiscale à l'article 265 du code des douanes dédiée au F10- indice 21 -, et de lui appliquer une taxe intérieure de consommation sur les produits ou TICPE, diminuée de 5 centimes d'euro par litre par rapport à celle qui est appliquée au fioul standard. En dotant le F10 d'une fiscalité adaptée, cette mesure est cohérente avec la stratégie du Gouvernement, pour au moins trois raisons. Premièrement, elle facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs gouvernementaux puisque le F10 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Deuxièmement, elle permettra d'atteindre un double objectif parfaitement cohérent avec l'ambition d'une neutralité carbone à l'horizon de 2050. En effet, en soutenant une incorporation plus grande des esters méthyliques d'acide gras, ou EMAG, cette mesure permettra d'offrir aux consommateurs- le plus souvent confrontés à des problématiques de précarité énergétique

en droite ligne avec les objectifs du Gouvernement, puisque le F10 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Ne nous privons pas de cette opportunité un nouveau produit qui permet de développer et d'atteindre de nouvelles stratégies pour les énergies nouvelles de demain. Le F10 est un nouveau type de fioul ayant vocation

n° I-199 rectifié. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, proche du précédent, cet amendement prévoit une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 30 % d'ester méthylique d'acides gras, ou EMAG, dit « F30 ». Il tend à créer une nouvelle ligne fiscale à l'article 265 du code des douanes pour le F30- indice 21 -et de lui appliquer un taux réduit de TICPE. En dotant le F30 d'une fiscalité adaptée, cette mesure est cohérente avec la stratégie du Gouvernement, pour au moins trois raisons. Premièrement, elle facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs gouvernementaux, puisque le F30 contribuera à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques. Plus généralement, cette mesure s'inscrit dans une perspective plus large de réduction de la consommation de fioul domestique. Deuxièmement, elle permettra d'atteindre un double objectif parfaitement cohérent avec l'ambition gouvernementale d'une neutralité carbone à l'horizon 2050. En effet, elle permettra notamment d'offrir aux consommateurs, le plus souvent confrontés à des problèmes de précarité énergétique, des alternatives crédibles et financièrement accessibles au fioul domestique 100 % fossile, ainsi que d'amorcer progressivement les évolutions nécessaires dans la perspective d'une sortie du fioul d'origine fossile à l'horizon 2050. Troisièmement, le F30 est un nouveau type de fioul ayant vocation à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul, avec le passage de 1 000 ppm à une obligation de 50 ppm prévue en France à l'horizon 2024.

produit à partir de colza. Sa distribution, encore progressive, a démarré en France dès le mois suivant dans plusieurs stations-service. Elle reste conditionnée, jusqu'en 2025, à la distribution, dans la même station-service, du carburant B7. Cet amendement est cohérent avec la stratégie gouvernementale, pour au moins trois raisons. En premier lieu, le développement du B10 participera pleinement à la transition énergétique, puisqu'il comporte une proportion accrue de biocarburants- à hauteur de 10 %. Il contribuera ainsi à la décarbonation du secteur des transports, qui restera encore largement dépendant des énergies fossiles dans les quinze prochaines années, conformément au scénario énergie-climat 2035-2050 de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. En deuxième lieu, la mesure vise à mettre en place une fiscalité incitative, qui permettra d'accompagner l'ensemble des Français dans la transition énergétique, tout en préservant leur pouvoir d'achat, dans un contexte où la hausse de la fiscalité sur les carburants pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages et provoque la colère des automobilistes, comme l'ont montré les importantes mobilisations de ces dernières semaines. En troisième lieu, ce dispositif participera à l'ambition affichée d'une fiscalité lisible, cohérente et non discriminatoire, puisqu'il permettra d'instaurer une égalité de traitement entre les filières essence et gazole. La Avec cet amendement, il est proposé d'appliquer au carburant B10 une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques diminuée de 2 centimes d'euro par litre par rapport à celle qui est appliquée au gazole standard, dit Le B10 est un carburant autorisé depuis juin 2018, qui contient jusqu'à 10 % de biodiesel produit à partir de colza. Sa distribution, encore progressive, a démarré en France dès le mois suivant dans plusieurs stations-service. Elle reste conditionnée à la distribution, dans la même station-service, du carburant B7 jusqu'en 2025. Cet amendement est cohérent avec la stratégie que prône actuellement le Gouvernement En outre, la mesure proposée vise à mettre en place une fiscalité incitative permettant d'accompagner l'ensemble des Français dans la transition énergétique, tout en préservant leur pouvoir d'achat, dans un contexte où la hausse de la fiscalité sur les carburants pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages.

qui ne sont pas concernés par les mesures de modulations locales ou de remboursements sectoriels. Tel est, par exemple, le cas du carburant B10, exclu du remboursement routier, du carburant B30, exclu du remboursement ferroviaire mis en place à l'article 19, ou encore du carburant E10, exclu du remboursement taxis. Ainsi, cet amendement prévoit que tous les carburants taxés comme le gazole ou l'essence, conformément au principe d'équivalence, c'est-à-dire à l'exclusion de ceux qui bénéficient d'un tarif spécifique, comme l'E85, de l'ED95 ou le B100, relèvent des dispositifs de remboursements ou de modulations locales. Cet amendement va dans le même sens que les trois amendements

Cette taxe est, en effet, basée sur le contenu carbone du gaz naturel, alors que le biométhane est un gaz vert produit à partir de déchets. Le montant de la TICPE appliquée au gaz naturel pour véhicules, le GNV, est aussi calculé à 100 % sur le contenu carbone de ce carburant. Cette taxe s'applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant, ou bioGNV. La valorisation du biométhane en carburant par l'utilisation du bioGNV est considérée par l'ADEME comme la plus vertueuse sur le plan environnemental. En l'état, elle deviendrait la plus taxée. Le présent amendement tend donc à prendre en compte le caractère renouvelable du bioGNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué. Sur le plan fiscal, il est en effet possible de distinguer le bioGNV, même mélangé à du GNV, en s'appuyant sur le système des garanties d'origine. Le registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-3 du code de l'énergie permet, en effet, d'assurer la traçabilité du biométhane, donc d'associer, d'un côté, les quantités injectées sur les réseaux et, de l'autre, les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.

Pourtant, la rédaction actuelle de l'article 265 du code des douanes pourrait être interprétée dans un sens contraire. Le présent amendement vise donc à en clarifier la rédaction, afin d'inscrire de façon claire et précise dans la loi l'exonération de TICPE voulue par le législateur, en complétant l'indice

M. Roland Courteau. À travers cet amendement, nous proposons que la trajectoire carbone qui a été fixée en juillet 2017 soit revue à la baisse.

si bien que la valeur de la tonne carbone pourrait atteindre 160 euros en 2030, contre 100 euros pour la trajectoire initiale ! Nous proposons donc de réviser la trajectoire actuelle sur le court terme, pour tenir compte des probables nouvelles hausses du prix du pétrole et laisser le temps aux gouvernements, d'ici à 2030, de mieux répartir les efforts et de repenser les mesures d'accompagnement en faveur des ménages pénalisés. Si la fiscalité écologique ne doit pas être destinée à fournir des recettes supplémentaires au Gouvernement pour compenser les baisses d'impôts, notamment aux plus aisés, elle doit surtout être un outil nécessaire pour réorienter nos modes de consommation et de production, à condition qu'elle soit juste, donc socialement inclusive. être accompagnée de mesures en faveur des catégories modestes et des ménages pour lesquels la voiture est incontournable pour se rendre au travail ou qui sont captifs des énergies fossiles pour se chauffer. À cette condition, la taxe carbone sera bien ce qu'elle doit être : un outil incitant chacun à modifier ses comportements, et non un prélèvement supplémentaire sur les classes populaires servant à financer les baisses d'impôts des classes aisées,

carbone a été progressivement augmenté par les lois de finances et suit désormais, en adéquation avec une cible de 100 euros par tonne de CO2 en 2030 prévue par la loi de transition énergétique de 2015, une trajectoire d'augmentation accélérée jusqu'en 2022. Cette trajectoire d'augmentation, confirmée par le projet de loi de finances pour 2019, est fondamentale pour rééquilibrer la compétitivité des énergies renouvelables. L'article 1 de la loi du 17 août 2015 de transition énergétique, sur laquelle s'appuie l'augmentation de la composante carbone des TIC, prévoit l' « élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, produits, travaux ou revenus. » Dans ce contexte, il est proposé d'asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d'exclure de la composante carbone les produits et énergies issus de la biomasse. Inscrire dans la loi de finances le principe selon lequel la composante carbone des taxes intérieures de consommation est assise uniquement sur le contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis permet de lui donner une valeur normative.

TIC, prévoit l'« élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des des émissions de gaz à effet de serre », ce qui n'est pas neutre, « cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus. » C'est dans ce contexte que nous proposons cet amendement.

afin d'exclure de la composante carbone les produits et énergies issus de la biomasse. Cette modification semble logique, car c'est l'exploitation de ressources fossiles carbonées qui engendre des excès de dioxyde carbone. Il est donc nécessaire de distinguer les deux origines de carbone et d'exempter le contenu en dioxyde de carbone des produits issus de la biomasse de l'augmentation de la contribution climat-énergie. Le vote de cet amendement donnerait également un signal positif au secteur des énergies renouvelables.

Mise en place par la loi de finances pour 2014, la composante carbone des taxes intérieures de consommation, ou TIC, a pour objet de moduler la fiscalité des produits en fonction des émissions de CO2. Le taux de la composante carbone a été progressivement augmenté par les lois de finances et suit désormais, en adéquation avec une cible de 100 euros par tonne de CO2 en 2030 prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, une trajectoire d'augmentation accélérée jusqu'en 2022. d'augmentation, confirmée par le projet de loi de finances pour 2019, est fondamentale pour rééquilibrer la compétitivité des énergies renouvelables. Dans ce contexte, il est proposé d'asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d'exclure de la composante carbone les produits et énergies issus de la biomasse. Inscrire dans la loi de finances le principe selon lequel la composante carbone des taxes intérieures de consommation est assise

Tous ces arguments sont connus et il est peut-être inutile d'y revenir trop longuement à ce stade. Je veux simplement indiquer, et cela ne surprendra personne, que le Gouvernement est défavorable à l'intégralité des amendements, y compris à celui de la commission.

me peine terriblement. Nous avons la capacité, dans ce pays, de proposer des énergies qui vont améliorer les énergies traditionnelles. Nous avons la possibilité, au travers de cette amélioration, de rendre les carburants fossiles Nous avons la possibilité de créer de l'emploi et d'améliorer notre compétitivité énergétique. Or nous ne nous en donnons pas les moyens. Je vais naturellement me rallier à la position de la commission,

Au reste, l'ensemble des amendements proposés par la commission des finances vont dans ce sens. Il faut de la clarté et de la lisibilité. Nos compatriotes, certains sont très excités, demandent à être considérés. Cet amendement est un amendement de considération et d'écoute à leur égard. Il ne remet pas en cause l'avenir d'une énergie moins carbonée, mais il temporise. Et il est temps de temporiser parce nous écoutons. Voilà la sagesse du Sénat ! Elle devrait être plus souvent suivie. C'est pourquoi je soutiendrai évidemment l'amendement de M. le rapporteur général.

que notre amendement soit soumis au vote du Sénat, puisqu'il prévoyait d'abaisser la trajectoire de la taxe carbone, laquelle a été considérablement rehaussée par l'actuel gouvernement.

de véritables mesures d'accompagnement en faveur des ménages pour lesquels la voiture est incontournable pour se rendre au travail, ou qui sont captifs des énergies fossiles pour se chauffer.

d'orienter et d'adapter la fiscalité écologique en fonction de la hausse du prix du pétrole, ce que n'a pas été capable de faire l'actuel gouvernement il y a un mois, et tout en rendant socialement inclusive dans la durée la transition énergétique, ce que ne permet pas l'amendement de la commission des finances. Car, à délai de trois ans, que se passera-t-il ? Je rappelle, et mon collègue Claude Raynal s'exprimera sur ce point, que nous restons favorables à un moratoire qui ne doit pas être un arrêt définitif. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons

Que je sache, le Sénat est plutôt réputé pour être une assemblée qui fait un travail de fond, qui essaye d'être la plus constructive possible et, surtout, qui écoute et porte la voix des territoires et de leurs élus, voire même de leurs habitants L'an passé, parce que le Gouvernement était quelque peu en lévitation et marchait sur l'eau, vous n'avez pas pensé qu'il était utile d'écouter la forme de sagesse que nous prônions et à laquelle nous vous avions invités.

assez curieusement, punir certaines activités industrielles considérées comme philosophiquement néfastes. C'est particulièrement vrai de l'énergie électrique lorsqu'elle est produite par le nucléaire, qui a l'immense mérite de donner à la France cette position du pays le plus décarboné d'Europe sur ce terrain. Oui ! Mais, sans qu'on en comprenne les raisons, on en limite la part dans la production d'électricité.

émet moins de particules fines que les moteurs à essence. La transition énergétique mériterait donc d'être revue à l'aune de la compétence dont Mme Ségolène Royal n'a pas fait particulièrement preuve, puisqu'elle a choisi la facilité en allant dans le sens

produit par les véhicules diesel, et un bon CO2 produit, par exemple, par la SNCF qui, elle, ne paie pas la taxe carbone. Des Français, lorsqu'ils font leur plein d'essence, paient plus de 60 % de taxes, quand d'autres, lorsqu'ils ont la chance d'accéder à des transports en commun, reçoivent plus de 60 % de subventions. comprendrez à cet instant que cela mérite réflexion ! C'est la raison pour laquelle je voterai l'amendement n° I-166, qui ne règle rien sur le fond, mais qui a le mérite d'ouvrir un moratoire. Espérons que celui-ci aboutisse à la mise en valeur des conclusions, que je partage totalement,

approuvions la transition écologique et la nécessité d'avoir des énergies non carbonées. Évidemment, nous partageons entièrement

ne la mordez pas ... Vous avez là une occasion d'écouter la voix de la sagesse, la voix de la raison. Prenez cette main, car le Sénat, c'est le monde de la proximité. Et c'est une collègue de votre ancien monde qui vous le dit, cet ancien monde qui connaît la proximité, cet ancien monde qui a le sens des réalités du quotidien de nos compatriotes, cet ancien monde de la ruralité, cet ancien monde de la France d'en bas, cet ancien monde de la France de ceux qui ne sont rien. Prenez cette main, écoutez-nous, et sachez que, oui, la République est certainement en marche. Marcher, oui, mais, comme dirait Aimé Césaire, marcher au pas du peuple

Jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a abandonné une énergie. Je suis favorable à la transition énergétique et à la décarbonisation de notre industrie et de notre mode de vie. En revanche, il faut bien se rendre compte que ce défi est inédit. Quand on a découvert le charbon, on n'a pas abandonné le bois : il s'est ajouté. Quand on a découvert le pétrole et le gaz, on n'a abandonné ni le charbon ni le bois. Quand on a découvert l'énergie nucléaire, on n'a abandonné ni le pétrole, ni le bois, ni le charbon. Quand on a découvert l'éolien, on n'a pas abandonné toutes les énergies précédentes. On a travaillé avec l'ensemble de ces énergies

de façon violente dans son mode de vie quotidien et qu'elle n'a pas les moyens de trouver une alternative. C'est la raison pour laquelle il me semble que la proposition du rapporteur général peut être écoutée. La parole est à M. Alain Joyandet, pour explication

qu'elle vous permet d'équilibrer vos orientations budgétaires, sur lesquelles, à titre personnel, je ne suis pas du tout d'accord. La taxe carbone ne peut pas servir à financer votre déséquilibre budgétaire. Vous ne pouvez pas financer la baisse ou la suppression de la taxe d'habitation par la taxe carbone ; vous ne pouvez pas financer la disparition de l'ISF par la taxe carbone. Car, au fond, c'est ce que vous faites

est tout de même un acte de cohésion sociale majeur. Vous ne pouvez pas faire payer au plus grand nombre, et bien souvent aux plus modestes, un certain nombre d'exonérations fiscales qui bénéficient au plus petit nombre.

Ces derniers ne remettent pas forcément en question le principe d'une fiscalité écologique, mais la manière dont est opérée cette taxation, ce qui conduit à la faire manquer cruellement de lisibilité- cela a été dit par un certain nombre d'orateurs

devons absolument nous pencher sur le dossier pour donner de la lisibilité à ces mesures et assurer l'irréversibilité de la transition écologique, car nous sommes à à une période de l'histoire où l'on ne pourra plus jamais fonctionner comme on l'a fait jusqu'à présent. Si l'on veut obtenir une acceptabilité sociale de ces mesures, il faut absolument qu'elles se traduisent par une forme de justice fiscale. C'est ce qui s'est exprimé dans les manifestations : de « gilets jaunes », puisqu'il faut les appeler ainsi, ont le sentiment d'une injustice fiscale, soit parce qu'ils habitent dans des lieux où ils cumulent toutes les taxes, soit parce qu'ils appartiennent à des catégories sociales qui sont

Il est fondamental que la question soit traitée dans son entièreté. Nous allons prendre des décisions concernant les taxes sur l'essence : pour ma part, je crois nécessaire d'arrêter les hausses qui étaient prévues,

la précarité, des dépenses contraintes- je pense au logement qui, comme les transports, pèse de plus en plus sur nos concitoyens -, et de la difficulté d'accès à certains services publics qui finit par coûter cher en transports.

on propose une justice fiscale inversée : il s'agit d'une première dans notre histoire, puisque ce sont les classes populaires et moyennes qui doivent financer la politique fiscale injuste menée par le Gouvernement.

Tout le monde dit, sur l'ensemble des travées, qu'il faut refaire ce budget qui ne correspond pas du tout aux nécessités. On est d'accord, même si nos solutions peuvent varier. Si cette augmentation de la TICPE avait été décidée l'an dernier en même temps que la suppression de l'ISF, notre collègue Alain Joyandet, nos concitoyens auraient peut-être fait le rapprochement entre les 4 milliards d'euros manquants d'un côté, et les 4 milliards d'euros s'additionnant de l'autre au niveau de la pompe ... Il y a tout de même une narration dans cette histoire : on a bien choisi, en urgence, de supprimer l'ISF parce que les gros patrimoines souffraient à n'en plus finir et qu'il était urgent de les soulager de cette charge insupportable et, l'année suivante seulement, d'augmenter la TICPE de pratiquement 4 milliards d'euros, dont 82 % de la hausse décidée entre 2017 et 2019 iront dans les caisses de l'État, et non pas à la transition écologique- cela a été dit, mais il faut le répéter. Dans le même temps, les dépenses consacrées à l'écologie diminuent de plusieurs centaines de millions d'euros. Un graphique récent émanant du ministère de la transition écologique faisait apparaître que plus les ménages avaient un niveau de vie élevé, moins ils étaient pénalisés par la montée en puissance des taxes écologiques. Je vous donnerai un chiffre : les 10 % des Français les plus pauvres perdront 2 % de leur revenu annuel à l'horizon 2022,

j'imagine bien- plusieurs de mes collègues l'ont dit -que vous n'avez pas forcément d'éléments sur ce que doit dire le Président de la République. Ayant connu cette situation, je ne vous en fais pas grief. Simplement, nous débattons et c'est le Parlement qui vote l'impôt et les dépenses publiques. Effectivement ! Franchement, nous laisser dans la situation de parler pendant des heures sur un amendement que je voterai, monsieur le rapporteur général, mais qui finalement demain sera peut-être déjà antique, cela donne le sentiment que le respect du Gouvernement pour le Parlement est assez faible, pour ne pas dire totalement délétère ... Ah oui ! Monsieur le secrétaire d'État, soit vous avez le sentiment

sur l'article suivant relatif au GNR. Il est vrai que, dans l'état actuel, si vous deviez adopter l'amendement de la commission des finances, cela reviendrait à la position de l'année dernière, c'est-à-dire le maintien du tarif de TICPE de 2018,

différer l'impact de l'augmentation du gazole non routier. Nous voulons très clairement en rester à la position que nous avions adoptée l'année dernière, c'est-à-dire le gel de la trajectoire,

d'être très variables, la position de clarté du Sénat, c'est d'en rester à notre position de l'année dernière : nous ne pouvons pas accepter cette hausse brutale sans accompagnement des Français. Je

dans les amendements qui ont été déposés. Aujourd'hui, les amendements intègrent le méthane dans le champ des exonérations, ce qui ne nous paraît pas opportun. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons le retrait des amendements, en prenant l'engagement- vous l'aurez compris au travers de mes propos antérieurs -de travailler sur ce sujet pour aboutir, notamment sur la question des biogaz.

les choses, et l'idée de le sous-amender ou de le laisser dans la navette me paraît assez opportune. Sinon, je crains de ne devoir le redéposer l'année prochaine, sans que cela ait vraiment évolué.

du prix du carburant et de l'énergie de chauffage, le présent amendement vise à instaurer un mécanisme permettant de préserver le pouvoir d'achat des ménages au moyen d'une TICPE flottante. La hausse du prix du pétrole ne doit pas permettre à l'État d'encaisser mécaniquement des recettes supplémentaires de TVA au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs- ménages et entreprises. Il convient par ailleurs de préciser qu'une forte proportion de l'augmentation récente des prix des carburants et du fioul domestique provenait de la matière première et, pour une part, de la fiscalité écologique. Par rapport à la hausse du prix du baril de pétrole,

En effet, si la TICPE est une taxe exprimée en euros, quel que soit le prix du pétrole,

dans les mois, voire dans les jours, à venir ; c'est comme si c'était écrit. D'où la proposition d'un mécanisme de TICPE flottante, qui permettrait, je le répète, de rendre aux consommateurs, sous forme d'une baisse de cette taxe, le surplus de TVA perçu. Un tel mécanisme avait d'ailleurs été mis en place en 2001. Quel est l'avis de

ici, peut nous assurer que le prix du baril ne va pas repartir à la hausse ? Faut-il ne rien faire, se contenter de dire « TICPE, TICPE ! » ? Dois-je rappeler la situation internationale, les problèmes du côté de l'Iran ou le fait que les États-Unis misent sur une hausse du cours du baril qui rendrait plus attractives, plus compétitives leur huile de gaz ou leur huile de schiste ? Ce que nous proposons, au travers de cet amendement, c'est d'anticiper une nouvelle flambée du prix du pétrole dans les semaines à venir, ce que le Gouvernement n'a pas su faire récemment

centimes, pour les ménages modestes, croyez-moi, ce ne serait pas dérisoire. Il faut, je le répète, anticiper toute hausse du prix du pétrole, car celle-ci, ajoutée à la hausse de la fiscalité écologique, peut être un coup de massue

qui peut accompagner l'évolution des cours du pétrole et adoucir un tant soit peu, dans certaines situations, les variations brutales des cours. La

il a permis d'éviter les dérapages de cours qui auraient eu un impact considérable sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est un outil de régulation, qui doit être utilisé quand il y a manifestement des abus du marché, qui fait des yoyo extrêmement importants. Je rappelle aussi que, quand on veut investir dans les économies d'énergie, mieux vaut avoir des prix de l'énergie relativement régulés plutôt que des hauts et des bas, parce qu'on sait qu'il existe des effets de dans les efforts que les uns ou les autres pourraient faire pour économiser l'énergie.

pour accompagner les ménages modestes dans la transition énergétique, en permettant à ces derniers d'obtenir des transferts fiscaux pour atténuer la perte de pouvoir d'achat provoquée par l'augmentation du coût du pétrole. Les mesures annoncées la semaine dernière par le Premier ministre ne sont pas de nature à convaincre nos concitoyens.

Cet amendement prévoit donc que des mesures supplémentaires soient mises en place pour venir en aide aux citoyens captifs de l'utilisation de la voiture, pour bonifier les aides à l'achat de voitures peu polluantes et lutter contre les « passoires énergétiques » en favorisant la rénovation des logements. La colère des Français qui s'exprime en ce moment au coeur du pays le vaut bien. Peu à peu, les raisons profondes de la démission de l'ancien ministre de la transition écologique se dévoilent. Le Gouvernement doit cesser de se réfugier dans une posture arrogante à l'égard de nos concitoyens et de nous enferrer dans une écologie punitive, qui met en danger la nécessité du consensus social le plus large possible.

au renforcement de la prime de conversion, sachant que personne n'imagine que cette prime permettra à tous les ménages français, en particulier à ceux qui sont le moins favorisés, de changer de véhicule, même si nous avons ouvert ce bénéfice aux voitures d'occasion récentes. Par ailleurs, le Gouvernement proposera,

qui ne fait qu'entretenir l'idée de l'injustice globale. Nos collègues socialistes ont raison d'essayer de limiter la casse, mais c'est quand même fondamentalement le principe de cette imposition

totalement injuste, inopérant, et que tous les bidouillages ne rattraperont pas ces injustices.

entre une station de distribution de carburant et la raffinerie la plus proche. En effet, la marge de distribution, qui est la différence entre le prix hors taxe à la pompe et le prix sorti de raffinerie, et qui ne désigne pas en tant que tel le profit du distributeur, est le prix payé par le consommateur pour rémunérer l'activité de transport et de distribution. Il résulte de cette situation un surcoût dommageable pour les usagers situés dans les territoires concernés, qui sont souvent des territoires ruraux et enclavés.

le taux de la TICPE, donc ce n'est pas tout à fait uniforme sur l'ensemble du territoire. Cela étant dit, quelle garantie aurait-on, si nous adoptions cet amendement, que le prix à la pompe baisserait véritablement

Les collectivités locales sont aujourd'hui les fers de lance de la transition énergétique, notamment par le biais de la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux à l'échelle des intercommunalités, par le biais du volet énergie des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires à l'échelle des régions, ou encore par la mise en oeuvre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Ces dispositifs doivent permettre de structurer la mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique. Néanmoins, le transfert de compétences envers les collectivités concernées n'a été accompagné d'aucun transfert de moyens. Cet amendement vise donc à attribuer une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités compétentes en matière de transition énergétique. Cette proposition a déjà été adoptée à deux reprises au Sénat, en 2016 et en 2017, par l'ensemble des groupes politiques. Elle est aujourd'hui soutenue par les territoires, par les structures représentatives des collectivités et par l'ensemble de nos concitoyens soucieux que l'action publique locale ait les moyens de ses ambitions en matière de transition énergétique.

sans pratiquement aucun transfert de moyens. Et sans moyens, ma crainte est que ces schémas ou plans ne soient pas pleinement mis en oeuvre, et ce d'autant que les restrictions budgétaires ne faciliteront pas la tâche. Or une grande partie des réponses de lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre se joue à l'échelle des collectivités.

l'amendement n° I-404 rectifié. Pour accompagner les territoires dans leurs investissements écologiques, cet amendement vise à créer des contrats territoriaux bas carboneentre l'État et les collectivités. Financés par une partie des recettes de la contribution climat-énergie, ou taxe carbone, ces contrats permettraient de fournir l'ingénierie nécessaire aux collectivités et donc d'enclencher, à court terme, ces projets d'avenir écologique. Nous touchons ici à un sujet essentiel. Comme vous le savez, monsieur le secrétaire la transition écologique passera d'abord par les territoires. L'expérience des territoires à énergie positive nous le démontre. Le récent rapport du GIEC relève, à maintes reprises, l'importance de l'action des territoires et des expériences locales pour concrétiser la lutte contre le réchauffement climatique. Cet amendement tend à traduire, d'une certaine manière, l'appel lancé en septembre dernier par le réseau CLER, qui fédère les territoires à énergie positive, ou TEPOS, pour que le Gouvernement accorde aux collectivités une plus grande confiance et des moyens pour passer à l'action. Ainsi, le fléchage d'une partie des recettes de la taxe carbone permettrait de viabiliser, sur le long terme, l'application des plans climat-air-énergie territoriaux, ainsi que les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADDET. de la cohérence en rendant aux acteurs de la transition énergétique les ressources financières apportées par la fiscalité écologique au lieu de les laisser abonder le budget général de l'État

qui, jusqu'à présent, n'étaient pas assurées par l'État, qui ne sont pas des transferts de compétences et qui, donc, ne relèvent pas du régime de transfert obligatoire des charges ainsi créées, faute d'être des charges transférées.

d'un projet de loi spécifique portant réforme de la fiscalité locale. Ce sera l'occasion de revoir l'affectation d'un certain nombre de produits d'impôts entre les différentes collectivités. Il nous paraît donc inopportun, à ce stade, de modifier la répartition du produit d'impôts nationaux en faveur des collectivités territoriales. J'ajoute, en écho aux propos de M. le rapporteur général, que les régions bénéficient déjà, au titre de leurs compétences, d'une fraction égale à 18

Vous vous souvenez de cette affaire : 22 milliards d'euros, puis 35 milliards d'euros ... Le compte n'y est pas et on va donc nous proposer d'alourdir encore une fois les taxes sur les entreprises, qui n'en peuvent plus et qui ont manifesté leur mécontentement. Peut-être, monsieur le secrétaire d'État, serait-il intelligent de regarder si une part de la TICPE prélevée en Île-de-France ne pourrait pas servir à financer la Société du Grand Paris qui construit ce supermétro ? Encore une fois, faire porter l'effort sur les entreprises me semble déraisonnable. Il y a des limites à tout. Notre collègue Dominati n'est pas là, mais je pense qu'il aura l'occasion de

je crois que ce gouvernement se caractérise par une nouvelle relation avec les collectivités territoriales, notamment sur le maintien de l'enveloppe globale des dotations. Arrêtez avec cette rengaine ! Madame la sénatrice, permettez-moi d'illustrer mon propos avec trois chiffres

l'annonce de suppression de ce dispositif a causé un grand émoi au sein des entreprises, notamment du BTP, qui dénoncent un coup de force du Gouvernement d'une brutalité certaine. certaine. Cette mesure n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les secteurs économiques concernés. En outre, elle n'aurait aucun caractère progressif, qui constitue pourtant un « principe de bonne politique fiscale pour donner de la visibilité aux acteurs ». Elle n'a pas non plus, semble-t-il, été évaluée sérieusement. Son impact direct serait de 500 millions d'euros pour la seule activité des travaux publics, soit environ 60 % de la marge des entreprises. Les entreprises du secteur, notamment, plaident pour une neutralisation des effets économiques de cette mesure, et elles évoquent, en cas de maintien en l'état, une déstabilisation certaine du secteur, particulièrement pour les PME. Nos entreprises du BTP en Martinique nous ont saisis sur le sujet, alors même que la TICPE n'est pas applicable dans les départements et territoires d'outre-mer, qui sont soumis à une taxe spéciale sur la consommation, la TSC, prévue par l'article 266 du code des douanes. Dans tous les cas, le taux de TSC retenu pour un produit ne peut excéder le taux de la taxe intérieure de consommation, la TIC, figurant au tableau B de l'article 265 du code des douanes. Or l'article 19 tend à opérer une modification de l'article 266 , dans la mesure où il réduit, sous couvert de simplification, la nomenclature des produits soumis à la taxe spéciale de consommation, ce qui fait disparaître l'alinéa relatif à l'« émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume » identifié à l'indice 53.

Cela équivaut, me semble-t-il, à une augmentation du taux de la taxe intérieure de consommation et, par conséquent, de la TSC. Étant de nature prudente et en l'absence de certitudes sur la réelle non-application de cette mesure dans nos territoires,

Cette mesure, socialement désastreuse, puisqu'on estime qu'elle ferait perdre en moyenne 313 euros par an à chaque foyer d'ici à 2022, ne saurait subir le verdissement ou de l'exécutif, lequel justifie cette hausse de la fiscalité carbone par une nécessité environnementale. Nous sommes dans le mensonge, nos débats de cet après-midi l'illustrent abondamment. Si le Gouvernement avait vraiment à coeur l'écologie et la bonne santé de la planète, il déploierait des alternatives aux transports individuels, Pascal Savoldelli vient de le dire. Il n'exonérerait pas fiscalement le kérosène pour les avions ni le fioul lourd pour les bateaux de croisière et les porte-containeurs. Enfin, il n'attribuerait pas seulement 19 % des recettes de cette fiscalité carbone à la transition énergétique. Notre Terre est malade. Notre population est toujours plus précarisée. Pendant que la maison France brûle, le Gouvernement regarde ailleurs, selon une formule ancienne, désormais célèbre, vers la seule réduction des déficits, dogme bruxellois par excellence. Les défis sociaux et environnementaux,

L'article 19 du projet de loi de finances est une disposition extrêmement importante, à savoir la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier. Le Gouvernement soutient, comme pour les autres augmentations de TICPE, que cette suppression est motivée par la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Néanmoins, notre collègue Maurice Antiste le disait il y a quelques instants, elle va déstabiliser très lourdement tout un secteur économique, en particulier le BTP, alors que, dans la plupart des cas, il n'existe pas d'alternative

absolument pas affectées à la transition écologique et à des modes de consommation plus durables. À preuve, selon les calculs du Gouvernement, cette suppression de tarifs réduits de GNR devrait rapporter 980 millions d'euros de recettes supplémentaires en 2019, ce qui s'ajoute aux 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires votés par la trajectoire carbone dans le projet de loi de finances pour

identiques, il s'agit de supprimer l'article 19, car ces dispositions ne peuvent que contribuer à grever lourdement les charges des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des carrières, qui sont utilisatrices de véhicules ou d'engins ayant recours à ce type de carburant. De nombreuses TPE du secteur du bâtiment ont une santé fragile, c'est peu de le dire, et cette mesure pénalisera nombre d'entre elles, alors même que le coût des carburants ne cesse d'augmenter, nous en avons parlé tout l'après-midi. Cette disposition est d'autant plus injuste qu'elle introduit une discrimination entre les entreprises du bâtiment, du paysage et des travaux publics

permet d'augmenter l'incitation à privilégier d'autres sources d'énergie que les énergies fossiles, dans le contexte de l'accélération de la transition énergétique ». Dans la mesure où, le plus souvent, il n'existe pas d'alternatives aux moteurs thermiques utilisés par les industriels, la suppression de cette dépense fiscale apparaît surtout comme une mesure de rendement.

paraît essentiel. Vous ne pouvez pas nous expliquer que vous maintenez les dotations des collectivités territoriales, que vous souhaitez que celles-ci fassent des efforts dans la gestion et, en même temps, au travers de cette disposition,

Cet alignement de la fiscalité du GNR sur celle du gazole engendrera pour les utilisateurs du GNR une hausse du prix du carburant de plus de 50 centimes par litre. Si les conséquences pour les TPE du bâtiment et des travaux publics, déjà fragilisées par la hausse continue du prix du carburant, seront considérables, cette suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR aura des conséquences pour nos collectivités. En particulier, les collectivités de montagne, au premier rang desquelles figurent les départements, assurent bien souvent le déneigement des routes à l'aide d'engins utilisant du GNR. Ainsi, pour le département des Hautes-Pyrénées, la suppression de tarif réduit de TICPE sur le GNR aura pour conséquence une hausse de l'ordre de 60 % du coût du carburant. Une telle augmentation viendrait une fois de plus rogner les budgets de nos collectivités, déjà soumis à nombre de baisses de ressources non compensées par l'État. Elle menacerait considérablement menacerait considérablement l'équilibre financier des stations de montagne. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

spécifique aux PME permettant de différer la mesure. Pour les plus grandes entreprises, je ne suis pas certain en effet qu'on puisse justifier qu'une très grande entreprise de travaux publics paye son carburant des dizaines de centimes de moins qu'un particulier. Dans ce cas, j'adhère à un mécanisme de répercussion, un mécanisme « pied de facture

Lorsque cette disposition a été adoptée à l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des finances s'est engagé à trouver des mesures visant à atténuer l'impact de la suppression du tarif réduit pour les secteurs les plus touchés, notamment les travaux publics et parmi les acteurs des travaux publics, les PME.

permettra, si vous l'adoptez, de limiter l'impact de la hausse du coût du GNR pour les contrats en cours dont la durée d'exécution est supérieure à trois mois. Par ailleurs, Bruno Le Maire avait annoncé une mesure de suramortissement permettant d'accompagner les secteurs consommateurs de GNR vers le renouvellement de leurs équipements, et nous travaillons actuellement sur la définition du champ de cette mesure. D'autres mesures sectorielles vous sont proposées. M. le rapporteur

Que, par ailleurs, on puisse solliciter, dans les grandes branches, des réflexions sur la mutation des outillages,

Les marges déjà réduites des distributeurs alimentaires qui utilisent des groupes frigorifiques seraient également fragilisées. Si les grands groupes devraient pouvoir absorber ce choc, il est en revanche à craindre que beaucoup de PME

Pour les raisons que j'ai déjà évoquées et que je veux bien répéter devant vous, la commission des finances considère que le problème se focalise d'abord sur les PME- le Gouvernement le reconnaît lui-même au travers de ses amendements -et, plutôt

! Nous sommes face à un gouvernement qui change d'avis ; ainsi, il annonce aujourd'hui qu'il va changer d'avis demain, après avoir indiqué très clairement qu'il ne changerait jamais d'avis

scrutin public, soient suivis avec passion par l'ensemble de l'opinion publique. En outre, nous risquons finalement d'être à contre-courant de ce que le Gouvernement va lui-même décider.

l'Assemblée nationale ne tiendra pas compte de notre position. Ce sera certes une satisfaction d'amour-propre pour ceux qui, comme moi, ont souhaité la suppression de cet article 19, mais nous n'aurons pas le débat auquel notre esprit de responsabilité nous a habitués. C'est pour cette seule raison que je vais suivre l'avis de mon groupe et refuser la

Comme pour la taxe carbone, le rapprochement de la fiscalité du diesel et de l'essence ou la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, une progressivité est nécessaire pour donner de la visibilité aux entreprises et leur permettre de s'adapter, par exemple en renouvelant leur parc de véhicules. Tel est l'objet de cet amendement. Les cinq

de type agricole ou forestier, comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles ayant au moins deux essieux, utilisés par des collectivités territoriales pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers, notamment le déneigement, continuent à bénéficier du taux réduit pour le GNR.

L'amendement a pour objet que les tracteurs de type agricole ou forestier, comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles ayant au moins deux essieux, utilisés par des collectivités territoriales pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers, notamment le déneigement, continuent à bénéficier du taux réduit pour le GNR. Si, au contraire, le taux réduit n'était plus appliqué pour le déneigement des routes, cela conduirait à une hausse du coût du carburant ; à titre d'exemple, pour le département des Hautes-Pyrénées, celle-ci Cette augmentation constituerait une ponction supplémentaire sur les budgets des départements, déjà lourdement obérés par une réduction continue de leurs ressources et une augmentation de leurs charges non compensées. L'effet cumulé des deux augmentations précitées, au total 50 centimes d'euros par litre d'ici au 1 janvier 2020, représenterait, pour le damage, 1 % du chiffre d'affaires, soit 20 % de la marge des entreprises, ce qui menacerait l'économie touristique des stations de montagne.

exemple le secteur agricole. Pour les secteurs économiques concernés- travaux publics, transports routiers, armateurs fluviaux, carrières ... -, cette mesure, applicable au 1 janvier 2019, est inacceptable, d'autant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable. Il convient également de noter que la suppression de cette exonération n'a aucun caractère progressif. Or les conséquences de cette hausse de la fiscalité seront effectives dès le 1 janvier 2019, alors même que tous les contrats en cours n'intègrent pas de clause de révision de prix, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. À titre d'exemple, dans le bâtiment, les contrats se font sur le long terme : une entreprise qui a signé un contrat au mois de septembre 2018 et qui ne réalisera le chantier qu'au mois de février 2019 devra assumer une charge supplémentaire. En conséquence, l'augmentation de la fiscalité ne pourra être répercutée sur le client et diminuera d'autant les marges des entreprises concernées. Il est à noter que les secteurs affectés ont de faibles marges et subissent une concurrence européenne et internationale importante.

L'alignement de la fiscalité du GNR sur celle du gazole va entraîner une hausse de près de 50 % du prix du carburant, qui sera difficilement imputable sur les clients, notamment les collectivités territoriales- comme

En outre, le phénomène des vols de carburant, auquel cette profession est malheureusement habituée, en sera certainement accentué. Il convient donc de maintenir le régime applicable existant. L'amendement n° I-1041, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances,

Cet amendement vise à proposer un dispositif alternatif en cas de maintien de l'article 19 du présent texte. Il tend à rendre éligibles les activités de déneigement des routes et d'entretien des pistes de ski au régime de remboursement applicable pour le gazole non routier des agriculteurs.

présenter l'amendement n° I-678 rectifié. Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier certains usages très spécifiques, aujourd'hui éligibles au gazole non routier, du même régime que celui mis en place pour les agriculteurs. Il s'agit des usages qui relèvent du service public et des missions de sécurité pour la gestion de la neige en montagne. L'exploitation des routes et des services publics est rendue plus complexe en montagne qu'en plaine par la présence de neige en période hivernale. Les surcoûts se traduisent notamment par le carburant nécessaire aux engins qui gèrent et déplacent la neige pour le bon fonctionnement des missions d'intérêt général et de service public, qui se déroulent sous le pouvoir de police du maire ou sous la responsabilité des départements. Le présent amendement tend à ne pas renforcer encore la pression sur ces collectivités de montagne, qui subissent depuis plusieurs années un effet de ciseaux sur leurs recettes et leurs dépenses. L'amendement vise l'ensemble des usages liés y compris ceux qui participent aux missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne telles que celles décrites à l'article 21 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

n'est pas soutenu.

Ces véhicules sont inclus dans la directive du 27 octobre 2003, qui fixe un cadre communautaire de taxation des produits énergétiques. Cet amendement tend à prendre en compte leur spécificité.

dans leurs véhicules, pour produire le froid nécessaire à la conservation des aliments jusqu'à leur lieu de distribution ou de consommation. Compte tenu des enjeux financiers pour les entreprises effectuant du transport routier de marchandises sous température dirigée et des effets induits, cet amendement a pour objet que le taux réduit de TICPE sur le GNR soit maintenu pour cette activité, dans l'intérêt économique, social et sanitaire de la France. Rappelons que ces mêmes entreprises sont par ailleurs soumises à de très lourdes incertitudes en matière de fiscalité foncière. liées à l'imprécision du régime de l'article 1499 du code général des impôts, conduisant les corps de contrôle à requalifier leurs entrepôts logistiques et de stockage en établissements industriels, avec, à la clé, des hausses de taxes pouvant dépasser les

amendement a pour objet de différer d'une année la hausse du tarif du gazole non routier pour le secteur du transport frigorifique, afin de permettre d'étudier un éventuel dispositif de répercussion des charges de gazole dans le prix appliqué pour leur prestation. Cette disposition sera mise en oeuvre une extension temporaire aux usages non routiers

de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, qui leur sont affectées. Il s'agit de tenir compte du décalage d'une année du remboursement ferroviaire, adopté à l'Assemblée nationale. Nous proposons les évolutions suivantes : tout d'abord, retirer les quantités de gazole non routier utilisées par le secteur ferroviaire en 2019 dans le calcul du coefficient de correction de cette année, afin de tenir compte du recours prolongé au gazole non routier par ce secteur ; ensuite, et c'est une nouvelle évolution, retenir pour le calcul du coefficient de correction les dernières quantités de gazole connues avant la réforme- celles qui ont été consommées en 2017 pour l'année 2019 et celles qui ont été consommées en 2018 pour les autres années -, en les corrigeant de l'estimation de la hausse des volumes jusqu'à l'année en cours.

de TICPE au 1 janvier 2019 ! Au sein de ces filières, pour les entreprises qui extraient et produisent des minéraux à usage industriel, un tel triplement serait extrêmement lourd de conséquences. La répercussion de la TICPE fragilisera les filières industrielles qui consomment ces minéraux à l'aval : industrie verrière, industrie céramique, industrie papetière, industrie forge, fonderie et métallurgie, Leur compétitivité sera directement affectée par rapport à leurs voisines européennes et internationales qui bénéficient de moindres coûts d'approvisionnement, d'énergies et de transformation- argiles d'Ukraine et de Turquie, talc australien et chinois, etc. Cet amendement vise, en conséquence, à prévoir un régime particulier pour les entreprises qui extraient et produisent des minéraux destinés à des applications industrielles, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les entreprises ferroviaires qui conserveront le tarif réduit en vigueur.

amendement vise, en conséquence, à prévoir un régime particulier pour les entreprises qui extraient et produisent des minéraux destinés à des applications industrielles, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les entreprises ferroviaires qui conserveront le tarif réduit en vigueur. Quel est l'avis de

Les dérogations autorisées par la directive et les règles communautaires ne concernent que des secteurs traités de manière nominative. L'agriculture et le secteur ferroviaire en font partie, ce qui préside aux amendements déposés à l'Assemblée nationale et à ceux que je défends devant vous ce soir. également de secteurs considérés comme extrêmement intensifs en matière énergétique. Tel est le cas du transport frigorifique, qui est considéré comme électro-intensif. Les industries extractives que les amendements déposés visent à faire sortir du champ de l'exonération

parlementaire et de constater qu'il y a des suppressions d'exonérations de gazole non routier proprement insupportables. Certains collègues ont évoqué les carrières.

explication de vote par l'exemple : dans mon département, une entreprise s'est adressée à moi pour m'indiquer que le surcroît de taxation

l'exemple type d'une mesure qui n'a pas été préparée et à laquelle les entreprises ne sont pas préparées. Encore une fois, ce qui est contestable, c'est sa brutalité. On ne peut pas, après avoir connu, durant des dizaines d'années, un différentiel de taxe,

vise à maintenir l'exonération de TICPE pour le gazole non routier utilisé par les entreprises de domaines skiables pour leurs opérations de damage. Nous souhaitons

de limiter l'impact de cette mesure pour les contrats en cours dont la durée d'exécution est supérieure à trois mois, dès lors que les entreprises concernées exercent des activités pour lesquelles l'utilisation du gazole non routier est significative, c'est-à-dire lorsqu'il représente en pratique au moins 2 % des coûts de production. Toutefois, seuls les contrats ne comportant pas de clause de révision des prix incluant le gazole non routier sont concernés. En effet, en l'absence d'une telle clause, les cocontractants ne peuvent pas ajuster le prix de leur contrat aux fluctuations des coûts de production. La préservation, pour ces entreprises, de l'équilibre économique résultant de ces contrats nécessite donc la mesure d'accompagnement contenue dans cet amendement.

Il en est de même s'agissant des entreprises appartenant au secteur de l'industrie extractive, que nous avons évoqué tout à l'heure. Pour rappel, le secteur des travaux publics en particulier est constitué à 98 % de TPE et de PME ; le taux de marge moyen est de l'ordre de 2 %. Pour certaines activités, le surcoût de gazole induit par la suppression du tarif réduit est donc potentiellement supérieur au résultat net de l'entreprise ; d'où cette mesure de précaution et d'accompagnement. La liste des activités concernées, ainsi que les coefficients de majoration destinés à prendre en compte l'impact de la différence de la fiscalité sur les coûts de production, seront fixés par arrêté et seront établis à partir des éléments statistiques de l'INSEE.

voter la suppression de cet article, nous n'en serions pas là et nous aurions rendu bien des services aux entreprises concernées,

Cet amendement vise à aménager un dispositif transitoire, afin de faciliter la distribution et l'utilisation du gazole coloré et tracé au cours de la première moitié de l'année 2019. Il est précisé qu'aucun rappel de taxes ne sera effectué auprès des utilisateurs de GNR pour les quantités de gazole acquises avant le 1 janvier 2019, mais utilisées entre cette date et le 1 avril 2019. De plus, une souplesse est aménagée pour les petits distributeurs de GNR. Ces derniers sont susceptibles de disposer d'une clientèle mixte, répartie entre le secteur agricole et les autres secteurs éligibles aujourd'hui au tarif réduit du GNR. La poursuite de l'approvisionnement de cette clientèle mixte nécessitera qu'ils disposent à terme de capacités de stockage et de capacités séparées pour le gazole coloré et tracé, taxé au tarif réduit, réservé aux usages agricoles, et pour le gazole traditionnel, taxé au tarif plein pour les autres usagers. Afin de laisser le temps nécessaire à ces évolutions, l'adoption de cet amendement aux distributeurs disposant de cuves pour un seul type de gazole de continuer, pendant six mois, à commercialiser du gazole coloré et tracé auprès de leur clientèle non agricole, sous réserve d'acquitter la différence de taxe entre le GNR et le gazole traditionnel auprès de la direction générale des douanes et droits indirects. Cette mesure vient en complément de la possibilité prévue au IV de l'article 19 pour tous les distributeurs de commercialiser du gazole non coloré et non tracé auprès des agriculteurs, puisque ces derniers bénéficient d'une procédure accélérée de remboursement.

En annonçant la suppression du taux réduit de la TICPE sur le gazole non routier, c'est une hausse d'impôts de près d'un milliard d'euros sur les entreprises que s'apprête à faire voter le Gouvernement.

Pour les 8 000 entreprises du secteur des travaux publics, dont 80 % sont des PME, cette hausse représente l'équivalent de 60 % de leur marge nette, dans un secteur qui se caractérise déjà par un faible taux de rentabilité nette- de l'ordre de 2 %. C'est une déstabilisation programmée du secteur, qui mettra en danger de nombreuses entreprises, en particulier les plus petites. L'impact de la suppression du taux réduit

La suppression de la réduction de la taxe sur le gazole non routier renchérirait les coûts de 3 % à 5 %, ce qui aurait nécessairement un impact sur le prix de sortie des logements et sur le volume de la commande publique. C'est pourquoi cet amendement vise,

Quel est l'avis de la commission ?

La loi fixe les plafonds des tarifs, qui ne peuvent pas être supérieurs à ceux qui sont applicables à la TICPE. Pour le reste, il appartient aux collectivités visées de prendre les délibérations qu'elle souhaite. Il revient donc à ces dernières, sous leur responsabilité, de modifier ou non la fiscalité sur le gazole non routier.

énergies fossiles pour amener à un changement de comportement. C'est absolument essentiel. Les seuls pays au monde qui tiennent les objectifs climat sont ceux qui taxent fortement le carbone-

d'autres termes, pour gagner quelques années de confort d'un monde qui ne change pas, c'est le monde de demain qui s'écroule. Cela ne marche pas. En revanche, et c'est là que le Gouvernement doit nous répondre, à partir du moment où l'on met en place ce type de taxation,

Sur l'ISF, dans la continuité de nos débats, je pense que votre groupe, comme le nôtre, présentera un amendement de rétablissement d'un impôt sur la fortune. Nul doute que la majorité sénatoriale y sera attentive ... Pour ce qui est de l'article

le rapporteur général.

Merci